La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur l'orientation des finances publiques et la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018 (projet n° 589, rapport n° 625). La conférence des présidents a décidé de joindre la discussion générale de ce projet de loi au débat sur l'orientation des finances publiques.

mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous retrouver- c'est désormais la troisième fois -pour ce débat d'orientation sur les finances publiques, qui nous donne l'occasion, à Gérald Darmanin et moi-même, de présenter les grandes orientations économiques et budgétaires du Gouvernement. Permettez-moi tout d'abord de faire un point sur la situation économique de la France. La croissance française reste solide malgré un ralentissement marqué et préoccupant de la croissance mondiale, lié en particulier aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. À ce stade, nous estimons notre croissance à 1,4 % en 2019, contre 1,3 % pour la zone euro et 0,8 % en Allemagne. Ces prévisions sont proches de celles des principaux instituts de conjoncture, ce qui confirme la sincérité à laquelle Gérald Darmanin

La conjoncture économique est inédite. Elle ouvre un cycle nouveau dans lequel l'inflation faible se conjugue avec une croissance mondiale faible et des taux d'intérêt durablement bas, voire même négatifs sur le court et moyen terme.

Cela étant, une croissance plus faible entraîne forcément une réduction des recettes fiscales, laquelle l'emporte sur la réduction de la charge de la dette. Par conséquent, il n'y a pas de cagnotte budgétaire liée à la diminution des taux d'intérêt.

doute un poison de plus en plus lent, mais cela reste toujours un poison. Nous sommes donc totalement déterminés à poursuivre le rétablissement de nos finances publiques et à réduire la dette française, même si nous assumons un niveau et un rythme de réduction plus lent, compte tenu de la situation conjoncturelle que je viens de décrire.

et l'emploi, en allégement de charges pérennes en 2019, pour 20 milliards d'euros, en est un premier signal très clair. Le deuxième signal, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner ce matin à cette même tribune, le taux de cet impôt sera porté pour toutes les entreprises, sans exception, à 25 % d'ici à 2022 et il baissera pour toutes les entreprises, sans exception, dès 2020. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros, le taux passera de 33,3 % à 31 %.

Aujourd'hui, la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Nous devons nous en réjouir et ne surtout pas changer de cap. Au total, les impôts baisseront de 13 milliards d'euros pour nos entreprises sur le quinquennat. Vous connaissez par ailleurs ma conviction quant à la poursuite de la réflexion que nous avons engagée ensemble au moment de l'adoption de la loi Pacte sur les impôts de production, qui, je le rappelle, sont beaucoup plus élevés en France que chez nos partenaires européens, et qui pénalisent en particulier les entreprises industrielles. Le pacte productif dont le Premier ministre et le Président de la République m'ont confié la mise en oeuvre sera l'occasion de faire des propositions sur le long terme sur les impôts de production.

Notre second choix économique, après la politique de l'offre, c'est la rémunération du travail. Le travail doit payer, et il doit payer mieux. La crise des gilets jaunes est pour moi une crise du travail,

La diminution de 5 milliards d'euros, pour 17 millions de Français, dès le 1 janvier 2020, de l'impôt sur le revenu s'inscrit exactement dans la même philosophie : le travail doit payer et les personnes qui ont un emploi doivent pouvoir vivre dignement de leur activité. Au total, ce sont 27 milliards d'euros d'impôts en moins pour les ménages sur l'ensemble du quinquennat, lesquels s'ajoutent aux 13 milliards d'euros de baisses d'impôts pour les entreprises, soit 40 milliards d'euros de diminutions d'impôts sur la durée du quinquennat. C'est l'une des baisses les plus importantes des dernières années, qui nous permet de rompre avec dix ans d'augmentation massive de la pression fiscale sur les entreprises comme sur les ménages. Quelles sont les conséquences en termes de finances publiques des choix que Gérald Darmanin Le rétablissement des finances publiques reste notre objectif et notre ligne stratégique. Le désendettement de la France, dont je viens de parler, est une nécessité à la fois pour notre bonne santé économique et pour notre indépendance politique de long terme. Le déficit public continuera de baisser. Il passera de 2,3 % hors CICE cette année à 2,1 % en 2020, soit nettement sous la barre des 3 %, que nous respectons depuis le début du quinquennat.

La suppression de ce tarif réduit permettra de dégager 900 millions d'euros à terme, un peu plus de 200 millions d'euros dès 2020. Par ailleurs, elle s'accompagnera de mesures de compensation qui ont été discutées avec les professionnels. Ainsi, nous mettrons en place une clause générale de révision des prix sur les contrats publics et privés

Le mécénat d'entreprise connaît une croissance extraordinairement dynamique : les dons et le nombre de mécènes sont en nette augmentation. Tant mieux ! Il n'est pas question de fragiliser cette dynamique, mais comme nous y invite le rapport publié l'année dernière par la Cour des comptes, certaines dérives doivent être corrigées.

La zone euro n'a pas vocation à vivre durablement avec une croissance faible. Il sera très difficile d'expliquer à nos concitoyens qu'elle est un succès,

Il est donc indispensable de réfléchir, en cette période de taux faible et dans l'environnement particulier que je vous ai décrit, à des moyens de relancer la croissance dans la zone euro.

Cette proposition me semble équitable, juste et responsable. Elle tient compte de l'environnement monétaire, beaucoup plus favorable, et de la baisse des taux d'intérêt. Elle prévoit d'avancer dans trois directions, en tenant compte des différences de situation qui existent entre les dix-neuf États membres de la zone euro.

depuis 2017 : le marché du travail, la formation, la qualification, la transformation fiscale, ou encore l'indemnisation du chômage. Le deuxième pilier, c'est le respect des engagements européens.

! Nous estimons qu'aujourd'hui l'Allemagne peut investir davantage dans ses infrastructures et dans l'innovation, pendant que la France poursuit le rétablissement de ses finances publiques et la transformation de son appareil productif grâce aux réformes de structure que nous avons engagées.

J'en suis d'autant plus heureux que les deux ne sont évidemment pas sans lien, le passé pouvant éclairer l'avenir. Le cycle budgétaire a d'ailleurs cela de rituel qu'il permet de traduire rapidement la volonté présidentielle et l'action du Gouvernement et de fournir, quelques mois après la nomination de celui-ci, un premier bilan. Comme le prouve le projet de loi de règlement des comptes, ce bilan est favorable, puisqu'il démontre que nous avons financé nos premières mesures en faveur du pouvoir d'achat, tout en étant sérieux budgétairement et en maîtrisant la dépense publique.

Notre devoir est de consolider les acquis du début du quinquennat et de poursuivre le rétablissement de nos comptes pour préserver la souveraineté budgétaire de notre pays, dont la signature est, comme vous l'aurez constaté, unanimement reconnue sur les marchés.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes en train de vivre un moment très particulier de notre histoire budgétaire et économique. Le 18 juin- date chère à la plupart d'entre nous -, la France a emprunté à des taux négatifs.

Depuis deux ans, le déficit est inférieur à 3 %, ce qui n'était jamais arrivé depuis dix ans. Comme le constate définitivement le projet de loi de règlement, le déficit des administrations publiques s'élève à 2,5 % contre un objectif de 2,7 % dans le dernier projet de loi de finances, soit une différence

Comme vous pouvez le constater, ce résultat est avant tout le fruit d'une meilleure maîtrise de la dépense publique qui a décru en volume en 2018 pour la première fois, mais aussi d'une budgétisation sincère et d'hypothèses macroéconomiques prudentes, comme l'ont souligné la Cour des comptes et le Haut Conseil des finances publiques. Le ratio de dépenses publiques rapportées au PIB est ainsi passé de 55 % à 54,4 % entre 2017 et 2018. Voilà plus de trente ans que cela n'était pas arrivé ! Dans les faits, les résultats sont là, et ce quels que soient les acteurs de la dépense publique.

Ces évolutions sont clairement en rupture avec les années passées, au cours desquelles la charge de la dette comme le budget européen étaient quasi systématiquement révisés à la baisse, ce qui facilitait l'exercice de bouclage du budget dans un contexte de dépassement budgétaire.

De fait, le redressement des comptes de la sécurité sociale s'est consolidé malgré le ralentissement conjoncturel du second semestre 2018 qui a pesé sur les recettes du régime général. Cela démontre qu'il est possible de tenir les comptes sociaux, désormais proches de l'équilibre- situation que la sécurité sociale n'a pas connue depuis 2001 -, tout en finançant les mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs. Dans les collectivités territoriales, mesdames, messieurs les sénateurs, force est de constater que la contractualisation, tant décriée, était conforme à la Constitution et qu'elle a bien fonctionné.

détail, sur l'ensemble du quinquennat, la croissance de la dépense publique en volume serait contenue à 0,2 % en moyenne contre 0,9 % sous le précédent quinquennat, alors même que nous avons rendu les dépenses de l'État sincères- plus de 7 milliards d'euros de crédits

cette séance à examiner à la fois le passé, en nous prononçant sur l'exécution de l'année 2018 et le respect de l'autorisation parlementaire issue de la loi de finances initiale, et l'avenir, avec le débat d'orientation de nos finances publiques pour 2020.

le déficit s'établit à 2,5 % en 2018, alors que le reste de la zone euro est à l'équilibre. Sur le plan de la dette, ce n'est pas mieux : le ratio d'endettement français est, pour la première fois, supérieur à celui du reste de la zone euro Le redressement nominal des comptes publics demeure porté par les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale qui confortent leurs excédents.

Encore une fois, les collectivités territoriales ont démontré leur capacité à participer à l'effort collectif de maîtrise de la dépense. Parallèlement à ces bons résultats des administrations locales, l'État voit, au contraire, son déficit se creuser de plus de 8 milliards d'euros par rapport à 2017,

Venons-en maintenant au débat d'orientation des finances publiques pour 2020. Comme l'an dernier, nous regrettons que cette étape de la procédure budgétaire n'apporte malheureusement pas beaucoup plus d'informations que le programme de stabilité en avril dernier,

Pour connaître ce que le Gouvernement souhaite faire, il vaut parfois mieux lire la presse, notamment la presse économique du matin, que les documents fournis à l'intention des parlementaires. Malgré de premiers chiffres plutôt décevants en 2019, le scénario de croissance, maintenu à 1,4 % pour la période 2019-2022, demeure crédible. La trajectoire budgétaire est encore davantage dégradée que dans le programme de stabilité, compte tenu de l'impact des mesures annoncées à la suite du grand débat national. Celles-ci ont un coût important, estimé à 6,4 milliards d'euros en 2020. Elles seront compensées à hauteur de 4 milliards d'euros. Non seulement

au début du quinquennat Hollande. Ce choix du Gouvernement de reporter le redressement des comptes publics marginalise encore un peu plus la France vis-à-vis de ses voisins. En commission des finances, très régulièrement, nous nous comparons à eux,

concentré sur les deux dernières années du quinquennat, ce qui paraît peu crédible. On n'a pas vu beaucoup de gouvernements engager des grandes mesures de réduction de la dépense à la veille d'élections.

En élargissant la perspective à l'ensemble des administrations de sécurité sociale, les ASSO comme l'on dit, l'excédent a augmenté en 2018 pour atteindre 10,8 milliards d'euros, soit 0,5 % du PIB. En citant ces chiffres, qui contrastent avec ce que nous avons pu entendre de la situation financière de l'État, nous pourrions croire que l'objectif tant attendu de retour à l'équilibre de la sécurité sociale est enfin atteint, et que le fameux « trou de la sécu » appartiendra bientôt au passé. je dois tempérer cet optimisme. Tout d'abord, parce que le résultat de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Cades, qui correspond au montant de la dette qu'elle a amortie l'année dernière, dépasse à lui tout seul l'excédent global des ASSO. Alors, certes, on peut considérer que, comme le dit l'adage, « qui paye ses dettes s'enrichit », mais, hors Cades, il est plus juste de parler de déficits amoindris que d'excédents dégagés par les ASSO. Ensuite, parce que l'amélioration des comptes de la sécurité sociale tient avant tout au fort dynamisme des recettes : hausse de 3,4 % en 2018 pour le régime général et le FSV,

le dynamisme d'autres recettes, comme les prélèvements sur les revenus patrimoniaux et les droits sur le tabac. En revanche, il faut relever que les dépenses de la sécurité sociale, soit 395,7 milliards d'euros pour le régime général et le FSV, ont, elles aussi, augmenté davantage que ce que nous avions prévu dans le cadre du PLFSS, et davantage que le PIB. La part des dépenses de la sécurité sociale dans la richesse nationale a donc continué de croître. Ne nous y trompons pas, la question du financement de la protection sociale reste un défi de long terme pour notre pays qu'un solde favorable une année donnée ne saurait masquer. Les principaux facteurs de croissance des dépenses sont bien connus. Il s'agit tout d'abord des dépenses maladie, même si l'Ondam a été respecté, au prix de réels efforts. Il s'est établi à 2,2 %, ce qui n'est pas négligeable en masse financière. Ensuite, les dépenses de retraite sont reparties à la hausse, 2,9 %, sous le double effet de la revalorisation de 0,8 % des pensions intervenue en octobre 2017 et de la fin des effets du recul progressif de l'âge de départ à la retraite.

Enfin, mon enthousiasme mesuré face à ces chiffres de 2018 tient évidemment aux perspectives de dégradation qui s'annoncent dès cette année. En effet, les prévisions de la commission des comptes de la sécurité sociale, confirmées par la Cour des comptes, sont pessimistes pour 2019. pour 2019. Ainsi, la croissance ralentit. La prévision du Gouvernement est désormais de 1,4 % en 2019, comme en 2020. Dès lors, la croissance de la masse salariale devrait, elle aussi, être moins forte. Dans le même temps, les dépenses poursuivront leur hausse, avec notamment un Ondam légèrement desserré. Ce seul effet croissance suffira à provoquer une légère rechute du « patient sécurité sociale » avec un déficit du régime général et du FSV qui se creuserait à 1,7 milliard d'euros sans mesure nouvelle. Cette rechute pourrait être beaucoup plus sérieuse en cas d'absence de compensation des mesures d'urgence économiques et sociales prises dans le cadre de la crise des gilets jaunes. Le déficit pourrait alors atteindre 4,4 milliards d'euros, effaçant presque les gains de 2018 et rendant plus complexes les perspectives de retour à l'équilibre. Dès lors, messieurs les ministres, je me tourne vers vous. Ce débat s'appelle « débat d'orientation des finances publiques ». Si les mots ont un sens, c'est le bon moment pour nous dire clairement vos intentions sur cette question importante de la compensation des mesures d'urgence. De quelles pertes de recettes pour la sécurité sociale liées à ces mesures proposerez-vous la compensation ou l'absence de compensation ?

le directeur de l'Acoss nous a dit lui-même que l'Agence, qui peut lever des fonds à taux négatif, allait une nouvelle fois être rémunérée pour emprunter, donc s'enrichir. Mais nous savons bien que céder à cette facilité ne serait pas de bonne politique et qu'il vaudrait mieux avoir traité la question de la dette le jour où les marchés se retourneront. Dans ces conditions, messieurs les ministres, pensez-vous qu'il sera possible de transférer une partie de la dette sociale actuellement supportée par l'Acoss à la Cades et, si oui, dans quelles conditions juridiques ? comme le Sénat l'avait dit dès l'année dernière, est-il bien raisonnable de mettre en oeuvre, à partir de 2020, les réductions successives de la part de TVA dévolue à la sécurité sociale prévues par la loi de finances pour 2019, en préemptant des excédents qui risquent de ne pas exister ? Là encore, ce débat me semble être le bon moment pour prendre une position claire sur cette question. Pour conclure, mes chers collègues, on pourrait dire que les comptes de la sécurité sociale ont connu une rémission en 2018. Hélas, une rechute est attendue pour cette année, mais sa gravité reste à déterminer. Elle dépendra pour partie des choix que nous ferons lors de l'examen des prochains textes financiers cet automne. J'informe le Sénat financiers cet automne. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget

Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, avec l'examen du projet de loi de règlement, nous achevons le cycle budgétaire tel qu'il est prévu par la LOLF. En constatant l'exécution budgétaire, cette étude permet aux parlementaires d'examiner les comptes de l'État et, plus encore, d'évaluer la performance de la loi de finances initiale. Nous débattons donc aujourd'hui non pas d'un simple document comptable, mais d'un vrai outil d'évaluation des politiques publiques, dans l'esprit des rédacteurs de la LOLF. Le projet de loi de règlement, que la commission des finances a adopté, présente les chiffres clés des finances publiques de notre pays : déficit, taux d'endettement, poids des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires. En 2017, le déficit est passé, pour la première fois depuis dix ans, sous la barre des 3 % du PIB. Rappelons-nous du contexte : ce résultat a été obtenu avec un effort en dépenses de 5 milliards d'euros et le remplacement de la taxe à 3 % censurée par le Conseil constitutionnel pour 5 milliards En 2018, le déficit s'est établi à 2,5 %. Il s'est de nouveau réduit, et davantage que la prévision retenue en loi de finances initiale. Le déficit public est ainsi amélioré de 0,3 point de PIB par rapport à cette prévision. L'endettement est L'endettement est quant à lui stabilisé, et la charge de la dette diminue légèrement grâce aux faibles taux d'intérêt. Le poids des dépenses publiques baisse de 0,6 point, atteignant 54,4 Le taux de prélèvements obligatoires diminue quant à lui de 0,2 point, et s'établit en 2018 à 45 % du produit intérieur brut. Ces chiffres, mes chers collègues, valident des choix de politique publique attendus par tous, élus comme citoyens. La baisse de la pression fiscale est une réalité. Je crois que nous pouvons dire qu'il s'agit d'une demande urgente des Français. La baisse du ratio de dépenses publiques dans le PIB crédibilise l'objectif d'une baisse de 3 points sur le quinquennat. Ces choix permettent des

Je le dis clairement, ces choix ont permis à l'économie française de créer de la richesse. Autre constatation, qui doit, au-delà de nos différences politiques, nous rassembler les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales sont en progression, notamment les dotations d'investissement, qui atteignent 1,482 milliard d'euros, et progressent de 409 millions d'euros par rapport à 2017. Cela est pour beaucoup dans la progression des investissements des collectivités territoriales territoriales de près de 8 % en 2018. Le FCTVA a augmenté de 510 millions d'euros l'an dernier. Je rappellerai l'élargissement de l'assiette aux dépenses de fonctionnement et d'entretien des bâtiments publics et de la voirie. Enfin, et avant la réforme de la fiscalité locale, qui nous occupera à partir de la rentrée, la TVA versée aux régions a augmenté. Ainsi, celles-ci sont largement bénéficiaires du remplacement de l'ancienne DGF des régions. Je veux faire un parallèle avec la réforme à venir à la suite de la suppression de la taxe d'habitation. Nous le savons, le scénario privilégié est l'affectation d'une part de TVA aux départements, avec la descente des taxes foncières de propriété au bloc communal. Selon ce scénario,

pour les départements en matière de recettes, mais nous devrons rester vigilants quant aux modalités pratiques de la réforme. Nous devons aussi collectivement souligner la bonne gestion budgétaire que révèle ce projet de loi de règlement. Je dis « collectivement », car la bonne adéquation entre autorisation en loi de finances initiale et exécution révélée en loi de règlement signifie que le pouvoir d'autorisation du Parlement a été respecté. Le taux de mise en réserve a été baissé de 8 % à 3 %, et il n'y a pas eu de décret d'avance en 2018, comme l'a souligné M. le finances. Par ailleurs, la publication du projet de loi de règlement a été avancée. Mes chers collègues, je conclurai mon intervention en m'exprimant brièvement sur l'orientation des finances publiques, c'est-à-dire le premier moment budgétaire de l'année 2020. Ce débat a lieu malgré les incertitudes autour des grandes données économiques. En effet, il n'est pas aisé de voir précisément où se situe l'économie française dans le cycle. L'inflation serait à 1,3 % en 2019, à 1,2 % selon les derniers chiffres de l'Insee. Il est difficile de dire, dans ces conditions, qu'il y a surchauffe. Il est Il est évident qu'il y a débat, et nous l'avons ici, sur le niveau d'endettement de notre pays. Je me réfère à l'article d'Olivier Blanchard de février dernier. Faut-il pour autant se réjouir que la France emprunte à taux négatif sur dix ans ? Je crois que cela pose davantage de questions que cela n'apporte de réponses, notamment sur les moyens de politique macroéconomique à notre disposition en cas de choc. Enfin, débattre sur l'orientation des finances publiques signifie débattre sur les choix.

plus présents sur les territoires ; cet équilibre demande, enfin, des baisses de la pression fiscale. À la suite du grand débat, le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé des mesures, que nous avons saluées : la baisse de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 5 milliards d'euros ; la reconduction de la prime exceptionnelle de fin d'année ; la réindexation des pensions inférieures à 2 000 euros mensuels. Ces mesures, évaluées à 6,4 milliards d'euros, doivent être financées grâce à un effort accru de maîtrise de la dépense publique et par la révision

consistant à vérifier la bonne exécution du budget de l'année antérieure. C'est surtout, selon nous, l'occasion de jauger l'efficacité et la pertinence des choix budgétaires faits par le Gouvernement. Au cours temps de parole- six minutes -qui m'est imparti, je n'entrerai pas dans le détail des recettes et des dépenses de la loi de finances pour 2018. Je me bornerai donc à évoquer quelques faits et constats saillants de cet exercice. Je souhaite d'abord revenir sur la suppression de l'ISF, décision idéologique très emblématique de ce gouvernement. L'un des arguments justifiant ce choix était de dire que la France était le seul État du monde à appliquer cet impôt. Or, curieusement, un débat sur ce sujet a lieu aux États-Unis en ce moment même.

Il est évidemment un peu tôt pour évaluer les effets de ce choix, mais il est d'ores et déjà possible de relever ici et là quelques indications. Deux sondages réalisés auprès d'anciens redevables de l'ISF confirment que l'élan vertueux espéré au service de l'économie productive se fait attendre.

Très grande sécheresse du côté du ruissellement escompté donc. Un économiste du MIT de Boston, évaluant les effets de la suppression des impôts sur la fortune dans d'autres pays que la France, à savoir le Danemark depuis 1996, l'Allemagne depuis 1997, la Suède depuis 2007, déclare : « Il n'y a aucune démonstration d'un effet visible et traçable sur l'économie ». Quelque chose me dit que le débat sur ce sujet n'est pas définitivement enterré, monsieur le ministre. Une loi de finances, un budget, est un outil indispensable pour garantir à chacun de nos concitoyens l'accès aux droits fondamentaux ; un outil, aussi, pour atténuer les inégalités criantes rongeant notre société, créant créant une situation d'injustice sociale qui a été relevée de manière spectaculaire depuis novembre dernier sur nos ronds-points et dans les rues de nos villes. La pauvreté sévit dans notre pays et les inégalités s'y aggravent. Citons les constats établis dans le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités en moyenne, les 10 % des Français les plus aisés perçoivent des revenus 8,7 fois supérieurs à ceux des 10 % les plus pauvres après impôts et prestations sociales. Notre pays est, après la Suisse- excusez du peu !-, le pays d'Europe où les riches sont les plus riches. En bas de l'échelle, 5 millions de personnes pauvres vivent avec moins de 855 euros par mois. Franchement, ce n'est pas la prime d'activité concédée au mouvement social qui va résorber ces écarts. Un mot, à ce stade, sur le choix de mettre en place le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU, la bien nommée. Cette décision a été l'un des piliers de la politique du Gouvernement. Le PFU de 30 % sur les revenus du capital n'a pas pesé sur le budget en raison d'une envolée des dividendes distribués en 2018. Notre pays, de ce point de vue, est devenu champion d'Europe L'augmentation de versement des dividendes a atteint 24,34 % en un an, à hauteur de 37,11 milliards d'euros. À l'évidence, les entreprises ont décidé de verser davantage de dividendes pour profiter d'une aubaine fiscale. De fait, le Gouvernement a subventionné le transfert des richesses vers les classes les plus élevées de la population. Vous appliquez le vieil adage libéral « trop d'impôt tue l'impôt », l'idée étant qu'un taux d'imposition bas peut rapporter au moins autant qu'un taux important, dans la mesure où la pression fiscale a des effets désincitatifs sur l'activité. C'est la fameuse courbe de Laffer, chère aux spécialistes. Cette théorie n'a jamais fait la preuve de sa pertinence. Si ! Les nombreuses expériences de baisses d'impôts, aux États-Unis comme ailleurs, en France notamment, ne se sont jamais traduites par une augmentation des recettes fiscales, bien au contraire. Elles ont davantage contribué à dégrader les comptes publics, sans compter l'effet des niches fiscales, qui permettent aux plus riches d'échapper à l'impôt. Messieurs les ministres, les baisses d'impôts et de cotisations ont un revers : elles affaiblissent singulièrement le système de redistribution et mettent la pression sur le budget de l'État. Au titre du bilan de l'année 2018, il conviendra aussi d'ajouter au passif la diminution des recettes du contrôle fiscal pour la troisième année consécutive. Les sommes notifiées par le fisc ont effectivement chuté, passant de 17,9 milliards d'euros en 2017 à 15,2 milliards en 2018. On apprend également, dans un article du journal du 20 juin dernier, que le fisc a abandonné un redressement de 1,4 milliard d'euros adressé La lutte contre la fraude fiscale ne fut pas évoquée un seul instant dans le discours de politique générale de M. le Premier ministre, prononcé à cette tribune, voilà quelques semaines. Ce silence ne manque pas d'interroger sur la volonté de ce gouvernement de s'attaquer de la plus forte des manières à ce scandale de notre temps. L'idée de création de l'Observatoire de la fraude fiscale garde toute sa pertinence. Faisons en sorte qu'elle ne disparaisse pas dans les limbes du renoncement et des influences. Ces résultats budgétaires ne sont pour nous en rien une surprise. Ils découlent mécaniquement des choix budgétaires et fiscaux que nous avions combattus lors du débat sur la loi de finances pour Ils ne prennent pas en compte la réalité économique et sociale de notre pays. Je citerai, pour conclure, les propos que M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État, a tenus dans une interview récente : « Il Il faut aussi avoir une vision claire du rôle de l'État dans la période actuelle de globalisation économique, de défis environnementaux et de fracturation de nos sociétés. Face à ces enjeux, l'État n'a jamais été autant concurrencé, subordonné, fragmenté, banalisé et paupérisé. Et pourtant, il reste ce qui fait que la société tient debout et ensemble. C'est le socle sur lequel la Nation s'est construite, dans un monde où les souverainetés sont battues en brèche par des entreprises multinationales qui se jouent des frontières ». L'État a été victime de la doxa libérale ». Cette doxa, messieurs les ministres, nous ne la partageons pas, et c'est donc fort logiquement que le groupe CRCE votera contre le projet de loi de règlement 2018. La parole

Il conduit à se pencher, d'une part, sur le passé, l'exécution effective des crédits, d'autre part, sur les projections pour les années à venir. Expression de la volonté d'une approche pluriannuelle de gestion des finances publiques, il éclaire particulièrement bien, à l'échelle d'un quinquennat, les choix politiques opérés par une majorité présidentielle. Je commencerai, si vous le voulez bien, par évoquer le projet de loi de règlement pour l'année 2018. Il convient, d'abord, de noter quelques points positifs en termes de pilotage budgétaire, liés notamment à la fin du recours à des décrets d'avance et à l'amélioration de la prévision budgétaire, ce qui se traduit par un recul des sous-budgétisations.

En premier lieu, notons la plus-value de 8,8 milliards d'euros de recettes fiscales par rapport à la prévision initiale, qui ne découle en rien de l'action du Gouvernement, mais dont nous ne pouvons que nous satisfaire. En second lieu, nous pouvons constater, voire dénoncer

du projet de loi de règlement pour 2017, vous nous aviez expliqué qu'en la matière, tout était de la faute du gouvernement précédent et que cela ne résultait pas de vos décisions politiques. C'est vrai ! Je suis curieux d'entendre cette année votre justification

destinés aux publics les plus fragiles a des conséquences sociales très claires. La montée en puissance des parcours emplois compétences, les PEC, qui ont remplacé les contrats aidés, reste inférieure à celle qui était prévue en loi de finances. En ce qui concerne les plans d'investissement dans les compétences, les PIC, 72,4 % des crédits de paiement ont été consommés, alors que vous aviez été alerté sur l'insuffisance de l'accompagnement prévu pour consommer efficacement ces crédits, pourtant fort utiles à leurs bénéficiaires.

exemples -, les conséquences de votre politique qui a conduit à une diminution de l'effort fiscal pour les plus aisés et à l'annonce d'actions non financées. Vous êtes amené, pour équilibrer vos comptes, à rogner sur des dépenses votées, sans apporter d'ailleurs aucune justification satisfaisante en la matière. Au-delà de cette méthodologie budgétaire, qui n'est pas sans interroger, vous vous targuez de résultats meilleurs que ceux de vos prédécesseurs, monsieur le ministre. Le déficit du budget de l'État est cependant resté très élevé l'an dernier. Il excède de 33,4 milliards d'euros le niveau qui permettrait de stabiliser la dette exprimée en points de PIB. Alors que, sous le quinquennat Hollande, la charge de la dette était passée au second rang des dépenses de l'État, elle repasse, cette année, au premier rang,

Nous vous avons également invité à « muscler » votre taxe sur les services numériques, qui reste à un niveau de rendement très faible. Nous vous avons suggéré, à de multiples reprises, de contenir le poids des niches fiscales. Comme l'a souligné le rapporteur général de notre commission des finances, elles ont continué à largement augmenter au titre de 2018. 2018. Rien n'y fait à ce jour ! Pour autant, je veux faire preuve d'optimisme et je me dis que mieux vaut tard que jamais. Du moins est-ce le message que je vous adresse aujourd'hui, monsieur le ministre. le ministre. En effet, vous semblez, de toute évidence, dans l'incapacité d'engager des réformes structurelles pour contenir le poids de la dépense publique, du moins sans pénaliser les personnes qui ont besoin du soutien de la puissance publique. Votre politique consiste à aider les multinationales, soutenir les grandes fortunes et équilibrer les comptes de la Nation sur le dos des plus faibles. Ce n'est pas acceptable ! Contrairement à vos affirmations toujours très positives, la publication par l'Insee des comptes de la Nation pour 2018 permet d'avoir une approche beaucoup plus nuancée clair, la politique du Gouvernement ne produit pas les résultats escomptés ! La croissance a été de 1,7 % en 2018, en recul par rapport à l'année précédente. La consommation contribue moins à la croissance qu'en 2017, avec 0,7 point. Enfin, le taux de marge des sociétés non financières décroît également. Si l'on ajoute à cela le retour à un accroissement des inégalités, on ne peut que conclure que la politique conduite par le Gouvernement est injuste sur le plan social et inefficace sur le plan économique. L'Insee met par ailleurs en avant le fait que, globalement, le seul secteur tirant véritablement son épingle du jeu en 2018 est celui des sociétés financières, dont l'activité se redresse. L'expression « président des très riches » qui fut accolée au Président de la République est donc aujourd'hui toujours d'actualité. Vous vous en doutez bien, mes chers collègues, d'une part, du fait de ces résultats économiques, d'autre part, en raison de la méthode consistant à sous-consommer des crédits pour équilibrer le budget, le groupe socialiste et républicain votera contre ce projet de loi de règlement pour 2018 Je veux enfin, mes chers collègues, évoquer rapidement le rapport préparatoire au débat d'orientation budgétaire. Malgré tous les indicateurs que je viens d'évoquer, le Gouvernement et votre ministère semblent considérer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est vrai, c'est indéniable, que la baisse des taux vous donne des marges de manoeuvre supplémentaires. Cependant,

Aujourd'hui, vous annoncez que le déficit public sera ramené à 1,2 % du PIB en fin de quinquennat et que la dette sera maintenue autour de 97 %. En juillet 2017, ici même, vous disiez : « Ces engagements sont chiffrés, monsieur le rapporteur général, vous pourrez le vérifier à la fin du mandat : faire baisser de trois points les dépenses publiques, de cinq points la dette et de deux points le déficit. Ces engagements sont extrêmement ambitieux. » Quelques mois plus tard, M. Le Maire, qui n'assiste plus à cette séance, indiquait : « Je souhaite à présent passer à un cap " l'objectif étant désormais de réduire la dette publique de huit points, pour qu'elle représente moins de 90 % du PIB en 2022. Je considère en effet que nous le devons à nos enfants et aux générations à venir.

Vous parlez de suppression de niches fiscales et de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État : c'est tout de même un peu léger, me semble-t-il. Un autre point mérite d'être évoqué, comme d'autres l'ont fait

le projet de loi de règlement que nous examinons aujourd'hui est le premier portant sur un budget voté et exécuté entièrement sous la nouvelle mandature. Le premier constat que l'on en tire est plutôt positif comme l'an passé, on constate une certaine amélioration des comptes de l'État. Le déficit effectif s'est réduit de 0,3 point par rapport à 2018, à 2,5 % du produit intérieur brut. Notre dette publique, pour la première fois depuis 2007, a cessé d'augmenter plus vite que notre PIB, s'établissant, comme l'année précédente, à 98,4 % du PIB. Cette embellie doit toutefois être tempérée par certains facteurs, mis au jour aussi bien par la Cour des comptes que par le rapport de notre collègue Albéric de Montgolfier. elle est en partie conjoncturelle, à la faveur d'une croissance plus forte que prévu, qui risque de s'essouffler dans les années à venir. D'autre part, elle ne permet pas de réduire l'écart qui sépare notre pays de la grande majorité de nos partenaires européens. L'assainissement de nos finances publiques doit donc se poursuivre, ce qui demandera de passer par des mesures structurelles. Nous pouvons, en ce moment, compter sur des taux d'intérêt très bas, voire parfois négatifs, mais nous devons garder à l'esprit que ces taux ne sont pas gravés dans le marbre. Notons toutefois que la trajectoire établie dans le projet de loi de finances pour 2019 a dû être corrigée à la baisse après les annonces intervenues en réponse au mouvement des « gilets jaunes Ces mesures ont ralenti l'effort de réduction de notre déficit. Il s'agit notamment de l'augmentation de la prime d'activité, de l'élargissement du chèque énergie, de la prime à la conversion ou encore de l'annulation de la hausse de la CSG pour les revenus les plus modestes. Je tiens pourtant à les saluer, tout du moins celles que je viens de citer, car elles vont dans le bon sens sur un sujet primordial : redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. C'est d'ailleurs là toute la difficulté, corréler l'équilibrage budgétaire et une amélioration du pouvoir d'achat des Français. La baisse des prélèvements obligatoires intervenue cette année doit être compensée. Reste à déterminer de quelle manière. Cela peut passer par une meilleure maîtrise de la dépense publique. Toutefois, attention à ne pas couper n'importe où Le Gouvernement semble avoir mis de côté le projet de suppression de 50 000 postes de fonctionnaires. Si tel est bien le cas, sans doute s'agit-il d'une sage décision. Il me semble en effet difficilement justifiable, dans un contexte de crise de l'éducation nationale et des hôpitaux, de réduire si massivement le nombre d'agents de la fonction publique, quand bien même les suppressions concerneraient d'autres domaines. Une autre solution, sur laquelle nous sommes tous d'accord, est d'encourager l'investissement. Or je me demande si les outils choisis jusqu'ici sont vraiment les bons. À commencer par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui a été pérennisé cette année en baisse de cotisations permanente. Rien ne permet de prouver que l'effort très important concédé par l'État soit amorti. On a beaucoup parlé- et on en parle encore aujourd'hui -de Conforama, qui ne constitue qu'un cas particulier, mais intéressant, à relever. L'entreprise s'apprête à supprimer 1 900 emplois en France. Elle a pourtant bénéficié de 63 millions d'euros de crédit d'impôt sur trois ans, dont l'utilisation peut poser question.

Peut-être devrions-nous envisager d'autres leviers en vue d'encourager l'investissement et de récupérer des milliards d'euros précieux pour notre équilibre budgétaire. Je tiens, par ailleurs, à souligner, après vous, monsieur le ministre, l'effort consenti par les collectivités territoriales. La progression de leurs dépenses de fonctionnement a été nettement moindre que l'objectif fixé dans le cadre de la contractualisation, se situant à 0,3 % contre une prévision de +1,2 %. se sont donc pleinement inscrites dans l'effort collectif de rationalisation des dépenses publiques. Les arbitrages ont sans doute été douloureux. Quoi qu'il en soit, les efforts consentis par les collectivités ont permis de dégager une marge de manoeuvre pour accroître les dépenses d'investissement, qui ont progressé de 4,9 % entre 2017 et 2018. Ce chiffre flatteur ne doit toutefois pas faire oublier la disparité des situations. Les territoires les plus fragiles doivent, plus que jamais, être accompagnés. Je pense réunir l'ensemble des élus du groupe du RDSE, dans toute sa diversité, en affirmant que nous devons mettre l'accent sur la fonction publique de proximité. Le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, a eu quelques mots encourageants pour les territoires. Il a dit vouloir « éviter de creuser un fossé entre deux France que certains voudraient opposer, mais qui ne peuvent ni vivre ni réussir l'une sans l'autre : la France des métropoles mondialisées et la France périphérique

Par ailleurs, la vitalité des territoires est irriguée par le tissu associatif, que certaines mesures ont mis à mal. Je pense à la suppression de l'impôt sur la fortune, qui a curieusement anesthésié la philanthropie des donateurs. Je pense également à la réduction du nombre de contrats aidés et, plus généralement, à la baisse notable des crédits de la mission « Travail et emploi ». Faisons très attention à ne pas abandonner nos associations ! En tant que rapporteur de la mission « Sport, jeunesse et solidarité », je serai particulièrement attentif aux conditions de la mise en place de l'Agence nationale du sport,

En 2018, les comptes sociaux se sont rapprochés de l'équilibre. Le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, est tombé à 1,2 milliard d'euros en 2018, contre 5 milliards d'euros en 2017. Les efforts doivent se poursuivre pour permettre à notre modèle social de fonctionner pleinement. Enfin, la Cour des comptes a relevé un effort de sincérisation du budget, que je ne peux que saluer. Il est primordial de se fonder sur des projections fiables afin de pouvoir maîtriser les dépenses. En conclusion, mes collègues du groupe du RDSE et moi-même voterons- avec quelques abstentions de règlement du budget et d'approbation des comptes, en espérant nous être fait entendre sur nos remarques. L'intérêt général et les services de proximité doivent être au coeur de nos réflexions budgétaires. Nos territoires ruraux ou périurbains, nos territoires d'outre-mer, nos petites villes et leurs habitants ne peuvent pas être oubliés. La parole

la discussion de ce jour sonne un peu comme une ode à Janus, le dieu aux deux visages : il s'agit de regarder à la fois le passé et le futur. C'est un peu ce que vous avez dit, monsieur le ministre. Le passé, afin de nous prononcer sur le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de 2018. Le futur, afin de débattre de l'orientation des finances publiques pour les années à venir. C'est aussi l'occasion de faire le point, à mi-mandat, sur la situation de nos finances publiques, de débattre de ce qui a été accompli, mais aussi, et surtout, de ce qui reste à accomplir. Ceux qui m'ont précédé à la tribune l'ont clairement dit, le Sénat continuera de se montrer exigeant pour poursuivre la diminution du déficit public et de la dépense publique. Toutefois, l'exigence n'interdit pas la bienveillance- et je dirais même que les deux vont plutôt bien ensemble. Le groupe Les Indépendants trouve dans les comptes de 2018 un motif de satisfaction, qui tient autant de la bienveillance que de l'exigence : nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons repris le contrôle de nos dépenses publiques. Et ce qui, outre-Rhin ou outre-Manche, relève déjà de l'évidence demeure en France un motif de réjouissance. Depuis trente ans, aucun gouvernement ni aucune majorité n'avait eu le courage et la rigueur de ramener le déficit public sous la barre des 3 % du PIB et de contenir l'augmentation de la dette publique. Ces bons résultats sont notamment dus aux excédents dégagés par les collectivités locales et la sécurité sociale, lesquels ont contribué à diminuer le déficit public en volume par rapport à 2017, et ce malgré l'augmentation du déficit budgétaire de l'État, qui, lui, s'est encore aggravé en 2018. Je tiens donc à saluer, au nom du groupe Les Indépendants, la contribution des collectivités territoriales à ces efforts budgétaires, notamment grâce aux quelque 5 milliards d'économies réalisées en 2018 sur leurs dépenses de fonctionnement.

C'est donc en grande partie grâce aux collectivités locales que le déficit public est passé, entre 2017 et 2018, de 2,8 % à 2,5 % du PIB. Mais cette bonne performance tient aussi et surtout à un fort dynamisme des recettes. La diminution du déficit nominal a ainsi été portée aux deux tiers par la conjoncture. Sur le même exercice, l'effort structurel n'a contribué à réduire le déficit qu'à hauteur de 0,1 point de PIB. C'est trop peu ! C'est trop peu, d'abord, car cela signifie que nous n'avons pas profité des temps cléments pour dégraisser l'État. C'est trop peu, ensuite, car notre pays fait encore figure, certains l'ont dit, de mauvais élève au sein de l'Union européenne. C'est trop peu, enfin, car cela signifie que nous devrons redoubler d'efforts à l'avenir, et ce dans un contexte politique et économique moins propice aux réformes structurelles. Vous m'accorderez que c'est rarement en juillet que l'on tient ses bonnes résolutions avec le plus de rigueur ! De même, c'est rarement à la fin d'un mandat que l'on tient ses bonnes résolutions ! À l'heure actuelle, la situation des finances publiques a cessé de se dégrader, qui est déjà en soi une bonne nouvelle, compte tenu de la pente sur laquelle notre pays était engagé, mais la situation ne s'améliore pas pour autant. Il nous faudra attendre 2022 pour espérer voir le poids de la dette diminuer par rapport à la richesse nationale. D'ici là, la dépense publique ne sera pas encore redescendue sous la barre symbolique des 50 % du PIB. Nous ne pouvons pas nous contenter de maîtriser la situation de nos finances publiques. La responsabilité nous oblige à les épurer, à les assainir. Il y a un an, presque jour pour jour, à cette même tribune, je partageais avec vous une conviction personnelle : l'histoire jugera ce quinquennat à l'aune de notre capacité collective à réduire notre dette. Je n'ai pas changé d'avis, et je continue de souhaiter la réussite de ce quinquennat. parce que nous pourrons ainsi redonner plus d'autonomie aux collectivités territoriales pour qu'elles s'affranchissent davantage de la tutelle de l'État. Parce que nous pourrons aussi regagner des marges de manoeuvre à l'échelle nationale pour assurer notre sécurité et gagner notre indépendance, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Parce que nous pourrons, enfin, ne pas laisser nos enfants payer le coût de notre manque collectif de courage. « Je ne remets jamais au lendemain ce que je peux faire le surlendemain », disait Oscar Wilde. Tâchons donc de ne pas suivre son exemple ! C'est pourquoi le groupe Les Indépendants votera en faveur du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes pour 2018, qui prend acte des efforts déjà réalisés. Nous continuerons également de soutenir, notamment lors de l'examen du budget à l'automne prochain, toutes les mesures qui permettront de poursuivre ces efforts dans la durée. La parole est à M. Vincent Delahaye.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que dire de ces comptes de 2018 ? Je résumerai ma pensée en ces termes : « Des progrès, mais peut mieux faire

Sur la sincérité, vous confirmez la rupture avec les pratiques de la précédente majorité socialiste consistant à ne pas inscrire dans le budget la totalité des dépenses futures.

Sur la prudence, en revanche, vos résultats sont moins réjouissants. Après trois années de stabilité relative, le montant du déficit, qui a nettement augmenté, est supérieur aux recettes de l'impôt sur le revenu. Cette situation est inquiétante, car elle est due au seul budget de l'État. Les collectivités locales sont en excédent, les administrations sociales aussi.

j'ai hâte de pouvoir vous présenter les nôtres, notamment la suppression de quatre-vingts niches fiscales. N'oublions pas la dette, qui s'élève à plus de 2 300 milliards Il faut bien avoir à l'esprit que le seul paiement des intérêts de la dette représente quand même l'équivalent du budget de la défense nationale ! Enfin, sur les économies, le compte n'y est pas. En 2018,

le nombre de fonctionnaires continue d'augmenter. On a malheureusement

vous devez impérativement baisser de façon significative la dépense publique. Baisser les impôts sans baisser la dépense, c'est une arnaque, dont le véritable nom est « impôt différé ». Il faut cesser de croire que la baisse de la dépense publique aurait des effets économiques négatifs. En matière de santé économique et budgétaire, comme en matière de santé physique, l'équilibre est la mère de toutes les vertus. raison pour laquelle l'équilibre budgétaire ne doit plus être un objectif, mais devenir une réalité. Et là, je ne suis pas optimiste ! Monsieur le ministre, au vu de tous ces éléments,

Le Sénat espère cependant qu'il s'agira du dernier où la Cour des comptes juge négativement les résultats de l'année passée, critiquant une « détérioration de la situation financière de l'État », ce que nous allons passer en revue. J'observe d'emblée que la dette française, contrairement à celle de la plupart des autres pays européens, ne diminue pas en 2018 et frôle même aujourd'hui les 100 % de la richesse nationale, ce qui pourrait, on le sait, poser de graves difficultés en cas de remontée des taux. Ma collègue Christine Lavarde y reviendra. Sur la forme, la Cour souligne, à juste raison, l'amélioration de la sincérité des comptes. S'agissant du taux de croissance économique, l'année 2018 a été, c'est également vrai, conforme aux prévisions avec une croissance de la richesse nationale de 1,7 %, qui accuse toutefois un ralentissement par rapport à 2017.

le Gouvernement a compensée en grande partie par la réduction du prélèvement sur recettes de l'État en faveur des collectivités locales. Je vous entends déjà me répondre, monsieur le ministre, que le déficit public s'est réduit de 0,3 point. Mais cette amélioration s'explique, notamment, par un excédent budgétaire des administrations de sécurité sociale- près de 11 milliards d'euros -et des administrations publiques locales- plus de 2 milliards d'euros -, ainsi que par une diminution de la charge de la dette rendue possible par la baisse des taux Cette amélioration repose par ailleurs essentiellement- et c'est ce qui est préoccupant -sur des facteurs conjoncturels, et non structurels, comme l'a d'ailleurs rappelé notre rapporteur général. le déficit public structurel, conséquence du report des réformes structurelles, ne diminue pratiquement pas en 2018. De surcroît, autre sujet d'inquiétude, la France demeure en queue du peloton des pays européens : la moitié de nos partenaires sont aujourd'hui en excédent budgétaire, et seules Chypre et la Roumanie ont un déficit supérieur à celui de la France, qui se trouve à égalité avec l'Espagne. Les dépenses de l'État ont continué d'augmenter en 2018, de près de 1 %, notamment en raison des hausses de dépenses de personnel. Celles-ci sont essentiellement dues aux recrutements de 2017 et à la montée en charge du protocole sur les parcours professionnels, carrières et rémunérations. Les dépenses des administrations de sécurité sociale ont également augmenté de 2,4 % en 2018, notamment les dépenses de la hausses ont été compensées par des recettes dynamiques. En revanche, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales ont été pour leur part maîtrisées, indépendamment du fait, d'ailleurs, qu'elles aient fait ou non l'objet d'une contractualisation.

près de 4 % pour les départements et de près de 2 % pour les régions. Côté recettes, en 2018, celles de l'État diminuent légèrement par rapport à 2017- une baisse de 1 milliard d'euros -en raison des allégements d'impôts. Les recettes fiscales du bloc communal continuent de progresser de 2,4 %. Cette progression est essentiellement due au dynamisme des bases. Les recettes fiscales des départements augmentent, elles, de 1 %, avec, d'ailleurs, une plus forte progression dans les départements peu peuplés.

ce qui pourrait inspirer le Gouvernement au moment de présenter son « acte III » de la décentralisation. En conclusion, monsieur le ministre- et je vous le dis très tranquillement -, il nous faut réformer l'État pour que celui-ci réponde mieux aux attentes des Français dans l'exercice des responsabilités qui sont les siennes, tout en dégageant de précieuses marges de manoeuvre budgétaires. Ces marges de manoeuvre sont nécessaires pour alléger le fardeau de la dette pesant sur la tête de chaque Français. de chaque Français. Elles sont indispensables pour permettre à la France de bien négocier le virage politique qu'elle entame, pour répondre aux défis écologiques, climatiques et environnementaux qui sont devant nous, et pour lesquels l'urgence à agir ne doit pas se confondre avec l'improvisation, la brutalité et la verticalité des annonces gouvernementales. Dans sa majorité, notre groupe votera contre ce projet de loi de règlement, mais certains d'entre nous choisiront de s'abstenir. La parole

le ministre de l'économie et des finances sur le mécénat, le CIR ou la détaxation du gazole ne se traduisent pas par une augmentation de la pression fiscale- en définitive,

Monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, une lecture rapide de l'évolution des ratios de la dette pourrait donner lieu à un satisfecit : pour la première fois depuis onze ans, la dette rapportée au PIB est stable, après une hausse de 0,7 point en 2017. En réalité, la situation patrimoniale de la France ne s'améliore pas. Malgré une augmentation des immobilisations sous l'effet de la revalorisation de l'indice des prix à la construction, la situation nette s'est encore dégradée de 33,7 milliards d'euros en 2018, sous l'effet de la hausse continue de la dette. Le besoin de financement de l'État a augmenté de 76 % depuis la crise de 2008. L'année 2018 ne déroge pas à la règle : 8,8 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires ont été mobilisés par rapport à 2017 pour couvrir principalement un déficit budgétaire de 8,3 milliards Une analyse de la Cour des comptes révèle que les déficits primaires cumulés sur la période allant de 2007 à 2018 expliquent, pour deux tiers, l'augmentation du ratio de la dette rapportée au PIB dans le cas français, contre moins d'un cinquième pour la zone euro. Nous n'arrivons pas à nous guérir du démon de la dépense publique Le montant de la dette cumulé a progressé de 56,6 milliards d'euros entre 2017 et 2018. À la fin de 2018, la dette des administrations publiques s'élève à 2 315,3 milliards d'euros. D'après l'Insee, ce montant s'établit à 2 358,9 milliards d'euros à la fin du premier trimestre de 2019, soit une augmentation de 43,6 milliards d'euros en trois mois

l'Ifrap, le maintien des taux à leur niveau de 2010 a permis à la France d'économiser près de 19 milliards d'euros entre 2010 et 2016 ; le Gouvernement annonce que 10 milliards d'euros supplémentaires seront économisés jusqu'en 2021. Cette situation conjoncturelle favorable ne doit pas nous rendre aveugles : une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nos têtes ! Selon les prévisions de l'Agence France Trésor, une augmentation des taux de 1

les conditions de financement favorables de la dette française par rapport à celles des autres pays de la zone euro ont masqué notre incapacité relative à réduire notre déficit structurel. Pour notre pays et pour les générations futures, nous espérons, comme le Gouvernement, que la croissance de la dette restera limitée en Nous constatons simplement qu'en un an le volontarisme a laissé place à une succession de dépenses budgétaires de court terme : alors que la réduction de la dette rapportée au PIB entre 2017 et 2022 devait être de 7,8 points dans le programme de stabilité d'avril 2018, contre 5 points prévus dans la loi de programmation des finances publiques, elle n'est plus que de 1,6 point dans le document d'orientation des finances publiques. Dans son rapport de janvier 2019, intitulé et réalisé à la demande de la commission des finances du Sénat, la Cour des comptes relève que « l'augmentation de la dette publique résulte en partie de l'absence de mécanismes contraignants de désendettement ». Monsieur le ministre, pourquoi ne pas copier les initiatives de la Suisse, de la Suède ou de l'Allemagne ? Le Parlement suisse a ainsi défini un frein à l'endettement, mécanisme budgétaire visant à éliminer le déficit structurel des finances fédérales. Le frein à l'endettement repose sur une règle simple : « sur l'ensemble d'un cycle conjoncturel, le montant total des dépenses ne doit pas excéder celui des recettes ». Dit autrement, dans ce paradigme budgétaire, seul un déficit conjoncturel est toléré. Ce mécanisme a fait ses preuves : en 2018, la Confédération suisse a dégagé un excédent de 2,9 milliards de francs suisses, après en avoir dégagé un de 4,8 milliards en 2017. Voilà qui laisse rêveur

Les objectifs que s'était donnés le gouvernement allemand en juillet 2015 à l'horizon de la fin de l'année 2019 seront tenus au-delà des espérances, puisque la dette publique est désormais inférieure à 60 % du PIB. Les exemples de nos voisins nous montrent que la dette n'est pas une fatalité

Par ailleurs, l'État devrait s'imposer à lui-même la règle d'or des collectivités locales : la section de fonctionnement doit s'équilibrer sans recours à l'emprunt ; l'endettement n'est pas mauvais en soi s'il sert à financer l'avenir. Le ministre Bruno Le Maire a invité l'Eurogroupe à signer un pacte de croissance, visant à profiter des taux d'intérêt bas pour avancer dans trois directions

est fait en matière de sincérité ; comme l'an passé, le déficit s'accroît ; comme l'an passé, les perspectives sont plus mauvaises

intervenant après une longue série d'orateurs dans cette discussion générale, je m'efforcerai d'allier concision et esprit de synthèse. Je me réjouis que nous examinions cet après-midi, tout à la fois, l'exécution des comptes de 2018 et les perspectives de nos finances publiques, selon le schéma vertueux qu'a voulu mettre en place le législateur organique, même s'il convient aussi de souligner les limites inhérentes à cet exercice annuel. Je reviendrai peu sur l'exécution de l'année passée, parce que le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux ont, chacun dans leur domaine, procédé à une analyse très approfondie de cette exécution budgétaire, notamment de sa conformité avec l'autorisation donnée donnée par le Parlement et avec les engagements du Gouvernement, qui figuraient également dans la loi de programmation des finances publiques. Leurs analyses sont détaillées dans deux tomes très documentés consacrés à l'exécution des comptes. Notre commission des finances a par ailleurs choisi, en plus des nombreux contrôles réalisés par les rapporteurs spéciaux, d'entendre plusieurs ministres sur les crédits de leur département ministériel, afin d'obtenir les éclairages nécessaires en vue de l'appréciation que nous pourrons porter, cet automne, sur le projet Globalement, l'exercice 2018 se caractérise par une meilleure sincérité budgétaire, même si des bémols peuvent être apportés, par exemple sur la manière dont on a utilisé ce que l'on nomme les « crédits non répartis

puisse nous dire si, oui ou non, il entend en tirer les conséquences dans une nouvelle loi de programmation des finances publiques, et à quelle échéance. Il nous appartient aussi, en qualité de parlementaires, de distinguer l'exercice purement comptable, qui peut être réussi, de l'évaluation de l'action publique. La sincérité mise en avant par le Gouvernement ne veut pas dire que le budget de 2018 fut un bon budget, et nombre d'entre nous s'étaient d'ailleurs opposés aux choix qu'il portait. Je pense en particulier aux coupes concernant le logement social ou les contrats aidés,

la LOLF, ne laisse aucune place à l'initiative parlementaire. L'absence totale du moindre amendement de séance aujourd'hui le démontre à l'évidence. En effet, son objet est simplement d'arrêter « le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle Elle concerne par ailleurs le seul budget de l'État, qui représente, je le rappelle, moins de 30 % de la dépense publique. Au minimum, une extension à l'exécution des comptes sociaux et des comptes locaux serait bienvenue, et les initiatives prises en ce domaine par la Cour des comptes vont dans le bon sens. La période de juillet devrait surtout être propice à une réflexion sur ce qui doit être fait en matière budgétaire et fiscale, compte tenu de la situation de nos comptes publics. Mais, comme chaque année, nous resterons sur notre faim, le Gouvernement ne donnant rien à voir réellement de ses intentions. Comme chaque année, les mesures fiscales seront dévoilées à l'automne, avec un temps très court pour que les acteurs, publics comme privés, puissent les analyser et s'y adapter. Nous l'avons vu l'an passé avec la mesure sur le gazole non routier par exemple. La ministre des transports vient certes d'annoncer la création d'une nouvelle taxe sur le transport aérien, mais l'information tombe au compte-gouttes et ne permet pas de disposer d'une vision d'ensemble. Je plaide, comme M. le rapporteur général, pour avancer le calendrier de la loi fiscale à l'été ; il serait possible ensuite de tirer les enseignements pour calibrer l'autorisation de dépense publique à l'automne.

sous l'impulsion du Président de la République, des baisses d'impôts d'un montant très significatif, répondant en partie aux demandes légitimes sur le pouvoir d'achat. Toute la difficulté est de savoir comment ces mesures, qui s'ajoutent à celles- déjà coûteuses -sur la taxe d'habitation, seront financées, dans un contexte où notre dette publique frôle les 100 % du PIB. Des efforts importants ont été engagés au cours des dernières années pour sortir la France de la procédure pour déficit excessif et, désormais, elle bénéficie d'un contexte économique et financier beaucoup plus favorable, avec des taux d'intérêt bas, voire négatifs. Cette situation confortable pour les décideurs publics ne doit pas anesthésier notre vigilance et la transformation de l'action publique reste nécessaire. Toutefois, cette transformation ne doit pas se faire au détriment des plus précaires, des plus fragiles, ni au service de quelques-uns Nous serons donc particulièrement attentifs aux dispositions proposées à l'automne, de même qu'à l'évaluation des mesures tant budgétaires que fiscales prises jusqu'à présent, notamment concernant l'imposition du patrimoine, sur laquelle, au sein de la commission des finances- M. le rapporteur général et moi-même

collègues,intervenant au nom du président Alain Milon, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des résultats et des perspectives financières des administrations de sécurité sociale : le rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe, l'a déjà très bien fait voilà quelques minutes. Je centrerai donc mon propos sur deux questions engageant les finances publiques et, plus particulièrement, les finances sociales : les retraites et l'assurance chômage. des retraites, comme Jean-Marie Vanlerenberghe l'a souligné dans sa présentation, les dépenses de la branche vieillesse sont reparties nettement à la hausse en 2018, de 2,9 % pour, environ, 134 milliards d'euros de prestations sur le seul régime général, et 236 milliards d'euros en comptant l'ensemble des régimes obligatoires de base. Cette hausse s'explique, d'une part, par l'effet en 2018 de la revalorisation des pensions de 0,8 % d'octobre 2017 et, d'autre part, par l'effet de la fin des mesures relatives à l'âge de départ. Sans nouvelle mesure, ce dernier effet va durer et la commission des comptes de la sécurité sociale s'attend à ce que le solde de la branche vieillesse replonge dans le rouge dès 2019. Face à ce constat, plusieurs choix sont possibles. On peut laisser filer les déficits, surtout en période de taux d'intérêt faibles, voire négatifs, mais cela n'est évidemment pas tenable à moyen terme. De plus, cela introduit un doute légitime, notamment parmi les jeunes générations, sur la viabilité de notre système par répartition. On peut rogner, année après année, le pouvoir d'achat des actuels retraités et reconnaissons, monsieur le ministre, que le Gouvernement a fait ce choix avec constance

quasi-gel de ces mêmes pensions en 2019, alors que l'inflation est repartie à la hausse, et la volonté affirmée de reconduire ce gel en 2020 pour, au moins, une fraction des retraités.

On peut enfin attaquer le problème à la racine et expliquer aux Français que les gains d'espérance de vie doivent se partager entre temps consacré au travail et temps passé en retraite.

Monsieur le ministre, au vu des sommes en jeu, il est légitime que vous expliquiez à la représentation nationale dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques ce que le Gouvernement proposera de faire cet automne pour équilibrer le système des retraites avant le passage à un système par points à l'horizon de 2025. S'agissant maintenant de l'assurance chômage, le Gouvernement a déjà dévoilé les grands axes de sa réforme, et notre commission a entendu Mme Pénicaud avant-hier à ce sujet.

En outre, ces modifications ne résolvent pas à elles seules le problème de la dette accumulée par l'Unédic, qui a atteint 35,3 milliards d'euros à la fin de 2018 et qui pourrait dépasser les 37 milliards d'euros à la fin de l'année en cours. Quelles sont donc les intentions du Gouvernement à l'égard de cette dette ? Compte-t-il laisser l'Unédic se débrouiller pour l'éponger, en comptant sur d'hypothétiques jours meilleurs ? Compte-t-il aider l'Unédic, en reprenant une partie de ses charges qui ne relèvent pas de manière évidente de ses missions, par exemple pour le financement de Pôle emploi ?

présentera ce texte ! Le débat commun est clos. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018.

Le scrutin est ouvert.

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace est parvenue à l'adoption d'un texte commun.